La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture.

les lois d’orientation sont élaborées pour répondre aux défis et aux enjeux spécifiques rencontrés par tel ou tel secteur. Or la première question que nous devons nous poser est de savoir si ce texte contribuera à ce que nos territoires puissent répondre aux demandes alimentaires des populations de demain. La décarbonation de notre agriculture, qui est la condition pour pérenniser le développement d’une agriculture nourricière tout en répondant aux défis climatiques, sera t elle suffisamment encouragée ? Le renouvellement des générations sera t il suffisamment soutenu ? La question du renouvellement des générations et de l’installation de jeunes en agriculture peut elle s’envisager sérieusement sans traiter la question du foncier ? C’est vraisemblablement pour éviter des querelles sur ce sujet que la question du foncier est très peu abordée dans ce texte. ce texte. Elle est pourtant centrale pour favoriser le renouvellement des générations, et la Safer pourrait ici jouer un rôle déterminant. Ce n’est pas une question secondaire. Comme le titrait récemment dans son éditorial un grand hebdomadaire national de l’agriculture, un montage sociétaire assez connu en France

Il n’y a pas si longtemps, près de chez nous, en Bretagne, il n’y avait de régisseur que celui qui régissait le domaine du château auquel était adossée une grande ferme. outre, toujours en matière de répartition des terres, il y aurait lieu de faciliter les échanges fonciers et de lever les obstacles aux échanges quand ceux ci résultent de qualifications différentes de l’usage des terres. Nous sommes en droit de douter, car ces questions sont centrales, plus encore dans une région comme la nôtre, la Bretagne, qui est d’abord une région d’élevage. Or nos élevages laitiers et bovins sont en souffrance

l’activité agricole est une activité humaine de production nourricière vitale pour le devenir de l’humanité. En second lieu, le fait d’avoir versé l’activité agricole dans la mondialisation des échanges et des prix conduit à des pertes de souveraineté dans le domaine alimentaire, car, quoi que l’on fasse, le poulet brésilien sera toujours moins cher à produire que le poulet de chez nous. Cela devrait donc nous inciter à rechercher de nouveaux dispositifs. S’il est vrai que les normes et autres contrôles tatillons ont de quoi exacerber les mécontentements, la chute de nos productions et les départs non compensés dans de nombreuses filières ont pour cause la rémunération insuffisante du travail paysan et son manque de lisibilité dans le temps. Ce n’est pas en renonçant à des ambitions agroécologiques visant à protéger la santé que nous garantirons l’avenir de notre agriculture.

Et pourtant, la question de fond devrait être celle du retour de la valeur ajoutée à la production, c’est à dire à la ferme. C’est cette course effrénée,

Les éléments sur la transition agroécologique et l’adaptation au changement climatique ont disparu du texte, alors que ces défis sont déterminants. La place accordée aux enjeux de revenus et de juste rémunération des agriculteurs, déjà faible initialement, a encore été réduite. L’ambition de renouvellement des générations, pourtant à l’origine de ce projet de loi, est considérablement amoindrie. Enfin, du point de vue de la souveraineté alimentaire, le texte aurait sans doute gagné à faire tant soit peu référence aux activités de pêche, qui participent aussi

Il aura au contraire des conséquences en cascade, souvent irréversibles, qui accroîtront la vulnérabilité du secteur. Ce sont là autant de raisons

Et si l’on ne fait rien, un tiers des fermes rescapées auront disparu d’ici à 2030. Cette alerte devrait à elle seule nous conduire à renverser la table. Le mal être est général. Qu’en est il donc de cette loi ? Après un parcours contrarié, la LOA arrive enfin jusqu’à nous, avec pour orientation très claire, hélas ! la fuite en avant. Ce texte aurait pu être l’occasion de s’engager avec détermination dans les changements systémiques qui s’imposent et d’entrevoir la possibilité d’un avenir meilleur. Mais il se complaît dans l’inaction coupable et risque même d’accélérer le processus de destruction du tissu agricole et rural. Une poursuite de la course mortifère, telle est la trajectoire choisie par les rapporteurs, avec comme seule boussole la compétitivité de l’agriculture et le triptyque « robotique, génétique, numérique » pour produire toujours plus ou, en réalité, pour limiter la baisse des rendements d’une agriculture qui altère les fertilités.

vous défendez une souveraineté stratégique qui se moque des droits individuels et collectifs, ici, comme à l’autre bout de la planète. De quelle souveraineté s’agit il donc ? Nous y reviendrons au cours des débats. produire, encore faut il savoir comment, quoi et pour qui. Devons nous produire en lâchant sur les normes et sur les droits, pour répondre à cette compétitivité internationale qui alimente le moins disant social et environnemental, ce modèle agricole qui détruit les conditions mêmes de sa survie, au profit de quelques gagnants temporaires à la tête des plus grosses industries agroalimentaires et au détriment de la majorité de nos agriculteurs Nous sommes également loin de l’ambition initiale du texte, qui devait apporter des solutions au défi du renouvellement des générations. Largement aggravé par le travail en commission, le résultat est caricatural. En vous acharnant contre toutes les solutions qui permettraient aux agriculteurs de devenir plus autonomes et de se passer des intrants chimiques, c’est notre souveraineté que vous attaquez. Quasiment toutes les références et les objectifs relatifs à l’agroécologie et à l’agriculture biologique ont été supprimés.

L’enseignement supérieur agricole devrait être un véritable outil stratégique de notre politique agricole. Vous préférez promouvoir un bachelor que la plupart des établissements n’ont pas les moyens de mettre en place. mais il n’y a toujours rien sur le revenu ! À peine cité dans l’article 1, le revenu digne est pourtant la demande principale du monde agricole – vous en avez parlé, monsieur le rapporteur. Le sujet sera t il traité un jour ?

Si la puissance publique n’agit pas pour renforcer la résilience de nos exploitations, le surcoût annuel lié à l’augmentation des aléas climatiques s’élèvera à 1 milliard d’euros, selon le Conseil

plus qu’aucune mesure contre les montages sociétaires, l’accaparement, la spéculation et la financiarisation. Existe t il vraiment une volonté de mettre fin à ce grand plan social en cours ? La question se pose légitimement. bio, alors que la filière subit la pire crise de son histoire, vous avez supprimé les objectifs chiffrés du texte initial : laissons faire le marché, notre santé passera après ! Nous sommes encore une fois dans une vision très aboutie des demandes de l’agrobusiness. Quelques mots sur l’installation

Enfin, nous souhaitons dénoncer les reculs en matière de droit de l’environnement, encore aggravés par le passage du texte en commission, notamment à l’article 13. En portant atteinte au droit de recours ou en ajoutant un critère d’intentionnalité presque impossible à prouver, dans les faits, vous dépénalisez la destruction d’espèces protégées. Cela constitue des régressions inédites. Désormais, c’est : des promoteurs immobiliers, énergéticiens et chasseurs malintentionnés – je n’inclus pas tout le monde – pourront détruire des espèces menacées et plaider la non intentionnalité, le tout sous couvert de « simplification administrative », bien évidemment. À ce projet déshumanisé, nous en opposons un autre : protéger et nourrir. Car telle est notre vision, celle d’une agriculture qui nourrit les humains et qui protège la terre et le vivant, soit l’assurance vie des agriculteurs. La prise en compte de l’ensemble des enjeux cités suppose une transition systémique. Cette transition agroécologique est non seulement un rêve, mais aussi une réalité efficiente, vécue par de très nombreux agriculteurs

Ceux qui voulaient que rien ne change sont satisfaits de cette loi. Mais nous ne lâcherons rien. Nous continuerons à relayer la voix des scientifiques et à accompagner les innovations des agriculteurs pour engager la nécessaire transition.

Nous allons donc examiner aujourd’hui la grande loi de programmation agricole, d’abord promesse de campagne du candidat Macron en 2022, puis promesse en réponse à la crise agricole du printemps 2024. Ce projet de loi d’orientation agricole se fonde sur trois constats implacables, dont tout d’abord celui d’une crise à la fois sanitaire et environnementale, ce qui va souvent de pair. Sur le plan sanitaire, la résurgence des épidémies d’influenza aviaire, de peste porcine africaine, de fièvre catarrhale ovine nous oblige à réfléchir à un meilleur accompagnement des filières en amont. Au niveau environnemental, le changement climatique met les facteurs de production sous pression : on le répète depuis longtemps déjà, et les conséquences sont de plus en plus visibles. Les rendements sont soumis aux aléas climatiques de manière croissante, que ce soit le gel, la grêle, le vent, la sécheresse ou encore les inondations. Je citerai en exemple l’année 2022, représentative du climat futur, selon Météo France, qui a vu les rendements des cultures d’été diminuer entre 4 % et 20 %. Toutes les projections scientifiques indiquent que la situation va encore se dégrader dans les prochaines années.

Autre constat, celui d’une crise économique et commerciale. Hausse des coûts de production, concurrence étrangère, relations commerciales tendues et, surtout, revenus insuffisants sont autant de raisons qui expliquent le mécontentement de tout un secteur. Si, d’un point de vue global, la France demeure largement souveraine en matière alimentaire et agricole, la situation est souvent contrastée selon les filières. Ainsi, le Haut Conseil pour le climat indique dans un rapport de janvier 2024 que « la France importe 20 % de son alimentation » et que ses importations alimentaires ont été multipliées par deux en valeur depuis 2000. Je pense au blé, au riz, aux viandes de volaille, aux fruits et légumes. Certaines limites se font jour et il convient d’assurer une réelle souveraineté alimentaire. Le troisième constat qui est aux prémices du projet de loi – il n’est pas de moindre importance – concerne la crise de renouvellement des générations. Le défi est de taille.

L’étude d’impact associée au projet de loi indique que « pour maintenir notre capacité à produire et à se nourrir, il serait nécessaire d’installer 20 000 agriculteurs par an, contre 15 000 actuellement ». Elle indique également que le déficit en actifs agricoles est d’ores et déjà très marqué, avec 70 000 postes à pouvoir. Ces trois constants sont alarmants. Nous ne pouvons qu’y souscrire. Ils expliquent en grande partie la colère légitime du monde agricole. Nous devons les garder en tête tout au long de nos débats, comme fil conducteur, et nous poser sans cesse cette question : comment y répondre ? L’idée d’une grande loi programmatique, censée pallier ces difficultés, est une idée louable. Je dis « censée », car les réponses proposées sont loin d’être à la hauteur, et en tant qu’ancien agriculteur, j’en suis le premier déçu. Telle qu’elle est rédigée, cette loi d’orientation agricole n’est que la prolongation de la politique libérale menée depuis de trop nombreuses années. Le texte est particulièrement imparfait pour deux raisons principales. Il l’est tout d’abord par son contenu. Nous aurons largement l’occasion d’en discuter, mais je souhaite aborder quelques points qui me paraissent essentiels. La portée de l’article 1 est par exemple difficile à saisir. Les notions de « potentiel agricole », d’« intérêt général majeur » et de « non régression de la souveraineté alimentaire » sont floues et sujettes à interprétation. Elles sous entendent en réalité une logique et elles pourraient à terme, notamment pour le principe de « non régression », participer à la remise en cause des réglementations environnementales. Ces formules incantatoires doivent être revues. Sur la notion de souveraineté alimentaire, je crois que nous passons complètement à côté de l’essentiel,

L’introduction, à l’article 13, du principe de « présomption de non intentionnalité » face à la destruction illicite d’habitats naturels ou de sites protégés me semble problématique et ressemble, à s’y méprendre, à un « permis de détruire la nature La Défenseure des droits s’est elle même montrée très critique vis à vis de l’article 15, qui vise à accélérer la prise de décision des juridictions en cas de contentieux contre des projets d’ouvrage hydraulique agricole. Cela conduirait à une restriction disproportionnée du droit au recours. 15, auxquels j’ajouterai l’article 17, constituent des régressions marquées en matière environnementale et nous proposerons de les supprimer en quasi totalité. Je précise, à titre

Je ne fais là qu’un constat… Mais, surtout, le projet de loi est imparfait au regard de toutes ses lacunes, de tous les manques et de toutes les thématiques restées sans réponse. Nombre de propositions cruciales qui constitueraient des réponses viables, concrètes et directes aux attentes des paysans ne sont pas évoquées dans le texte et seront considérées comme irrecevables durant nos discussions. aucune mesure sur le revenu agricole alors que, en trente ans, le revenu net de la branche agricole a baissé de près de 40 % en France en euros constants, avec une forte hétérogénéité en fonction des catégories d’exploitation. Les agriculteurs ne demandent qu’à vivre dignement de leur travail

Aucune mesure sur le foncier pour lutter contre l’accaparement des terres. Il s’agit pourtant d’un élément indispensable à l’installation de nouvelles exploitations. Nous ne pourrons pas faire l’économie d’une grande loi foncière. Aucune mesure de réorientation de la PAC, alors que nous savons très bien que 25 % des agriculteurs

nous qualifier, mes chers collègues : nous souhaitons simplement installer de jeunes agriculteurs sur des sols qui fonctionnent ; nous souhaitons simplement que l’exercice de leur métier ne les rende pas malades ; nous souhaitons simplement que les agriculteurs puissent produire une alimentation saine et accessible à tous ; nous souhaitons simplement permettre aux paysans de vivre de leur métier.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi d’orientation agricole n’est rien d’autre que la botte de paille de Gabriel Attal, il y a un an, ce jeune « bobo » parisien en costume cravate et chaussures Weston qui joue au paysan devant un parterre de journalistes sans apporter de réponses à la hauteur des enjeux. Depuis les manifestations de colère historiques de nos paysans en février 2024, aucune des trois grandes promesses n’a été tenue. Les importations d’Ukraine continuent d’inonder notre marché national. Des accords internationaux autres que le Mercosur, comme l’accord économique et commercial global (Ceta), sont toujours sur la table. Le pacte vert, pacte de décroissance et de corruption, avec ses 10 % de jachères et sa folie normative, est toujours là. Le moment de clarté imposé par Donald Trump doit nous conduire à sortir du moment de confusion macronien dans lequel tous les partis politiques qui ont soutenu la construction européenne et l’idéologie décroissante se retrouvent aujourd’hui. Toute promesse à l’égard de la ruralité et du travail paysan sera vaine si vous ne décidez pas de sortir de vos ambiguïtés structurelles. En effet, madame la ministre, vous ne pouvez pas parler de « souveraineté alimentaire et agricole » sans sortir des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). J’ai d’ailleurs déposé une proposition de loi constitutionnelle pour reconnaître cette exception agriculturelle. Il faut donc que vous préfériez nos paysans à l’OMC. Madame la ministre, vous ne pouvez pas encourager la concurrence libre et non faussée à l’intérieur de l’Union européenne tout en poursuivant le harcèlement bureaucratique et la surtransposition des directives européennes en matière agricole qui aggravent la concurrence déloyale. Pour réussir, il faut préférer nos paysans à la fausse morale décroissante.

Il faut donc préférer nos paysans à l’OFB, aux ONG et à l’Union européenne. Madame la ministre, vous ne pouvez pas participer à un exécutif qui soutient Ursula von der Leyen, la fédéraliste européenne, « en même temps » qu’il inscrit la souveraineté alimentaire et agricole dans la loi française. Vous devez définitivement préférer les paysans français à la à la Mère Fouettarde allemande ! Sans volonté d’avoir une action claire pour sortir de ces impasses, vous réduisez ce texte à un feu de paille porté par des hommes de paille et condamnant le reste de nos agriculteurs à finir… sur la paille ! L’agriculture française sera souveraine si les paysans vivent souverainement de leur travail et ont la capacité d’en transmettre le fruit sans être étouffés par la fiscalité, la souveraineté agricole et la dignité paysanne allant de pair. Madame la ministre, nous savons que, depuis le mois de juillet dernier, l’agenda du président Macron s’est considérablement allégé, au point de lui permettre de s’occuper des prix du billet d’entrée au Louvre ou du paiement du péage autoroutier avec un smartphone. Aussi,

Ces débats traînent depuis juin dernier, ce qui nous aura au moins permis d’avoir un peu plus de temps pour analyser la situation et choisir les combats prioritaires à mener. Nous sommes prêts aujourd’hui à en discuter et à faire de ce texte un nouveau moteur pour l’agriculture française. Cette réussite passe par des décisions claires, efficaces et, surtout, en adéquation avec les réalités auxquelles font face nos agriculteurs. Le regard des Français sur l’agriculture doit changer. Il est temps de stopper le des détracteurs de la ferme France. Nos agriculteurs souffrent, le métier n’attire plus, faute de rémunération suffisante. Les précédentes crises, notamment l’invasion de l’Ukraine, nous ont rappelé à quel point notre indépendance énergétique et alimentaire est aujourd’hui indispensable. Stop à la surréglementation, à l’inflation normative et à la surtransposition ! Notre agriculture doit retrouver son rang de premier exportateur européen. Je tiens à saluer la réactivité du gouvernement Attal, qui avait su apporter des réponses concrètes lors de la crise agricole de janvier 2024, notamment face à la maladie Depuis lors, les tensions se sont de nouveau exacerbées lors des négociations entre l’Europe et le Mercosur. Alors oui, des solutions conjoncturelles et rapides sont indispensables. C’est pourquoi je nous félicite d’avoir adopté la semaine dernière la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. C’est une réponse directe à certaines difficultés rencontrées par la profession. à quelques semaines du salon de l’agriculture, nous savons que les attentes sont aussi fortes que justifiées. Au delà des crises ponctuelles, la multiplicité des enjeux auxquels nous sommes collectivement confrontés appelle des solutions structurelles. Tel est l’objet de ce projet de loi. Il ne s’agit ni d’une loi d’urgence ni d’une loi de circonstance, mais d’un texte d’orientation, qui déterminera la direction que nous entendons donner à notre agriculture à l’avenir. assurer notre souveraineté alimentaire, la transmission et le renouvellement des générations. Ce projet de loi doit s’inscrire dans la durée comme une première étape de planification. Dans le contexte international actuel, nous devons nous demander si une nation incapable de produire ce qu’elle consomme peut encore espérer rester indépendante. Je tiens à saluer le travail réalisé sur ce texte par plusieurs de nos collègues députés pour enrichir certaines définitions et préciser des dispositions. Le projet de loi initial était déjà issu d’un long travail de contributions et de réflexion. Néanmoins, toutes les évolutions ne sont pas au niveau des enjeux, et le texte reste insatisfaisant en l’état. Je salue le premier travail effectué par mes collègues issus des différentes commissions saisies, notamment au sein de la commission des affaires économiques. Nos échanges nous permettront de simplifier certaines dispositions et d’en préciser d’autres. À l’article 1, les précisions apportées à l’Assemblée nationale, sous la houlette du groupe Horizons & Indépendants, étaient les plus susceptibles de répondre à ces défis. Largement réécrit en commission, cet article doit consacrer la souveraineté alimentaire,

les trop nombreuses cessations d’activité ne sont pas compensées. Malheureusement, le temps perdu ne se rattrape pas. Aussi, je vous propose d’employer celui qui nous reste avec une efficacité redoublée.

Les nouveaux exploitants ne veulent pas forcément être propriétaires de leurs terres, ou ne le peuvent simplement pas. Nous devons donc réfléchir à de nouveaux outils, et leur en proposer.

Nous aurons également l’occasion de revenir sur la haie, le défrichement et les installations d’assainissement. Le groupe Les Indépendants est, et restera, très investi et attentif durant nos échanges, qui s’annoncent longs et passionnés,

Les origines de ces crises sont bien connues. Entre les surtranspositions pénalisantes, une bureaucratie tatillonne, des règles de négociations commerciales trop peu respectées et mal sanctionnées, des accords de libre échange mortifères et un climat politico médiatique qui alimente l’agri , , comment s’étonner de l’effondrement de notre compétitivité et du découragement du monde paysan ? Notre agriculture est confrontée à des défis immenses, et je veux souligner ici le soutien inconditionnel et constant de la majorité sénatoriale au monde agricole. Le travail mené par les deux rapporteurs du texte que nous examinons aujourd’hui en est une nouvelle illustration. Comme l’a rappelé Laurent Duplomb, ce projet de loi d’orientation agricole porte assez mal son nom, tant il se montre trop bavard sur certains sujets et étonnamment muet sur d’autres. Les amendements adoptés en commission ont heureusement permis d’en corriger de nombreux aspects, d’en renforcer la normativité et d’en simplifier le contenu. Le Sénat a par exemple enrichi les dispositions en matière d’installation et de transmission des exploitations agricoles. Il y a urgence à agir quand on sait que, d’ici à 2030, la France pourrait perdre encore 47 000 exploitations et qu’un tiers des agriculteurs seront partis à la retraite. Je pourrais aussi citer toutes les dispositions permettant d’alléger les contraintes et la pression psychologique pesant sur les agriculteurs en cas de contrôle et de sanction, ou encore la réécriture complète de l’article sur le statut et le régime juridique des haies.

Chacun le sait, si ce projet de loi contient des avancées importantes, il ne produira pas non plus de miracle. Ce texte ne doit être que l’un des maillons d’une séquence agricole plus vaste, composée de textes parlementaires et de mesures budgétaires. Je pense en particulier à la réforme des retraites agricoles sur les vingt cinq meilleures années que nous défendons depuis longtemps au Sénat. Un nouveau mode de calcul est rendu nécessaire par l’aggravation des aléas climatiques et l’instabilité croissante des revenus des agriculteurs. Cette réforme entrera en vigueur dès le 1 janvier 2026, si et seulement si le projet de loi de financement de la sécurité sociale est adopté. Elle permettra d’augmenter la pension des polypensionnés et de rendre les travailleurs non salariés agricoles exerçant leur activité à titre secondaire éligibles aux minima de pension. J’en profite pour rappeler, madame la ministre, qu’il est indispensable que la rétroactivité, prévue à partir de mars 2028, ne soit appliquée que pour des cas très exceptionnels. La réponse à la crise agricole passe aussi par l’Union européenne, et l’on ne peut que regretter ici la perte d’influence de la France à Bruxelles, où notre voix ne porte plus. La résolution européenne sur la politique agricole commune adoptée par notre assemblée en décembre dernier montre que le chemin est encore long. Les solutions futures de la PAC seront cruciales pour la sécurité alimentaire et la stabilisation des revenus des agriculteurs. Pour conclure, mes chers collègues, l’agriculture est à un tournant de son histoire. Si nous ne réagissons pas maintenant, il sera bientôt trop tard. Défendre notre agriculture, ce n’est pas seulement défendre nos agriculteurs : c’est aussi défendre les Français et leur droit à une alimentation saine et sûre. Il s’agit aussi d’un enjeu de santé publique. Madame la ministre, nous vous attendons donc ici comme à Bruxelles ! Pour cette raison, et parce que les attentes sur le terrain n’ont jamais été aussi fortes, nous voterons en faveur de ce projet de loi. La parole

après plusieurs mois d’attente et de reports, l’examen de ce texte, quelques jours après l’adoption de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, est une excellente nouvelle. La vocation de ce texte, tant attendu par les acteurs du monde agricole, est double. D’une part, il s’agit de traiter les problématiques liées à l’orientation, à la formation, à la transmission et à l’installation. texte doit apporter des réponses concrètes à la mobilisation des agriculteurs qui a eu lieu au début de l’année 2024. Alors qu’un agriculteur sur deux aura atteint l’âge de la retraite d’ici à 2030, l’immense défi du renouvellement des générations est devant nous. Si ce projet de loi entérine la création d’un guichet unique d’accueil, d’orientation et d’accompagnement, dénommé France installations transmissions, chacun sait que cette seule mesure ne suffira pas. La crise démographique à l’œuvre dans le monde agricole n’est pas une fatalité. J’en veux pour exemple mon département, le Doubs, où l’agriculture est principalement orientée vers l’élevage bovin laitier. d’origine contrôlée (AOC), la population d’exploitants y est la plus jeune de France, avec un âge moyen avoisinant les 47 ans. Le taux de remplacement y est proche de 95 %, grâce à une bonne dynamique d’installation 80 à 100 installations par an. Mon territoire en est la preuve : le sujet de l’attractivité des métiers agricoles auprès des jeunes est intimement lié à celui de la viabilité du modèle économique des exploitations. Tout en s’adaptant aux multiples transitions qu’ils observent en première ligne, celles et ceux qui nous nourrissent doivent continuer d’assurer leur mission première. Nous soutenons l’initiative des rapporteurs d’introduire à l’article 1 un principe de non régression de la souveraineté alimentaire de la Nation. L’ambition de ce texte en matière de formation est louable tant l’enseignement agricole constitue un puissant levier pour transmettre aux jeunes générations les compétences d’aujourd’hui et de demain. La formation à l’agriculture biologique, financée à hauteur de 180 millions d’euros chaque année, ne doit pas être oubliée. Il serait contre productif et incohérent d’opposer les modèles. Plus largement, nous devons retisser des liens entre l’agriculture et notre société. J’ai la conviction que l’établissement du programme national d’orientation et de découverte des métiers agricoles, prévu par ce texte, y contribuera. consacré à la simplification normative. Il est urgent de faciliter la vie de nos agriculteurs, victimes de la complexité du cadre réglementaire et législatif qui leur est imposé. Si ce texte comporte bien quelques réponses en matière de gestion des haies ou d’approvisionnement en eau, il nous faudra aller beaucoup plus loin. Je veux dire un mot du devenir de la profession vétérinaire, dont chacun sait le rôle essentiel qu’elle joue dans le monde agricole. L’article 7 du projet de loi, travaillé avec les organisations professionnelles concernées, vise à autoriser les auxiliaires vétérinaires justifiant de compétences certifiées à réaliser certains actes de médecine et de chirurgie vétérinaires. Madame la ministre, afin de préserver le fruit d’un large compromis, nous comptons sur votre extrême vigilance pour que le décret d’application demeure fidèle au contenu de cet article. Enfin, sénatrice d’un territoire dont les éleveurs subissent la présence du loup, force est de constater que les dispositions prévues par l’article 16 n’auront qu’une portée limitée. Cette question devrait continuer à être traitée dans les prochaines années, car c’est bien l’avenir de l’élevage français qui est en jeu. Le projet de loi, sans résoudre tous les problèmes,

Madame la présidente, mes chers collègues, « vieux monde qui se meurt », « clair obscur d’où surgissent les monstres » : vous vous êtes inspirée, madame la ministre, de la pensée d’Antonio Gramsci,

En 2014, prenant acte de la nécessité et de l’urgence d’une action publique en faveur du climat et de l’environnement, la France se dotait d’une loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Cette loi portait sur les fonts baptismaux l’agroécologie, en lui fixant un triple objectif de performance économique, sociale et environnementale. Dix ans plus tard, une évaluation, ou du moins un point de situation au regard de ces objectifs, aurait été utile pour répondre aux difficultés identifiées et prolonger la démarche avec une efficacité accrue. En effet, sauf à considérer qu’il n’y a rien à faire et que les tendances observées doivent se poursuivre, certains sujets conditionnent fortement le devenir de l’agriculture française à l’ère des transitions écologique et énergétique. La diminution très forte du nombre d’exploitations et d’emplois, les difficultés à recruter du personnel, les pertes de surface utile ou encore le niveau des rémunérations illustrent le caractère darwinien des évolutions à l’œuvre. La sélection économique naturelle se poursuit inéluctablement Dans ce contexte, les expressions récentes et diverses de la profession agricole auraient mérité d’être mieux entendues et prises en compte pour répondre aux difficultés. Je pense en premier lieu à celles qui sont relatives au revenu. À partir d’une très bonne idée, celle des États généraux de l’alimentation, les lois Égalim se sont succédé sans apporter de solutions satisfaisantes ou pérennes aux agriculteurs les plus en difficulté. Tant que cette question ne sera pas résolue, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les agriculteurs manifesteront, à juste titre, et on trouvera de moins en moins de candidats à l’installation ou à la reprise… Rien, hélas ! dans le texte dont nous allons débattre ne nous permettra de leur apporter des solutions sur ce point. La formation, le conseil et le diagnostic des exploitations, au demeurant nécessaires et même développés à haut niveau, ne répondront pas à la question du revenu pour le plus grand nombre. Dans un contexte de concurrence souvent exacerbée où le marché fait loi, le développement de l’agroécologie nécessite aussi la définition et la mise en œuvre d’outils de régulation des marchés et des prix. Pourtant, des outils disponibles pourraient être mis en œuvre, comme le fonds de stabilisation du revenu agricole que le groupe socialiste avait fait adopter ici même en 2016 ; Henri Cabanel s’en souvient. La PAC actuelle contribue au revenu des agriculteurs, mais de façon uniforme et rigide. Sans pouvoir de marché – et c’est le cœur du problème –, les producteurs subissent d’autant plus la volatilité des prix que tous les mécanismes de régulation qui existaient ont disparu. Le dernier en date était celui des quotas laitiers. Sa suppression a entraîné à une nouvelle étape de réduction de la polyculture élevage sur certains territoires, comme dans le département du Gers. Dans l’Union européenne, peu de pays ont mis en place des dispositifs de gestion des risques de marché, alors que le règlement n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 le permet toujours. Il serait également utile de réfléchir à la régulation de certains marchés à partir de corridors de prix, entre prix plancher et prix plafond, comme c’est le cas dans d’autres secteurs économiques.

Plus fondamentalement, la question des modèles agricoles que les États membres entendent soutenir se pose. Dans l’objectif d’un approfondissement du modèle agroécologique et d’une meilleure prise en compte du travail des agriculteurs, la PAC devrait progressivement passer

que vous nous exposiez votre vision des évolutions souhaitables de la PAC pour soutenir le revenu du plus grand nombre d’agriculteurs dans un contexte de transition écologique qui reste à approfondir. Je pense tout particulièrement à la qualité biologique et sanitaire des sols et au maintien de la polyculture élevage, absolument vitale pour le devenir de pans entiers de notre territoire national. Il n’est pas trop tôt pour engager ce débat à propos de la prochaine PAC et du plan stratégique national de la France qui en résultera. Nous regrettons aussi que ce projet de loi ne contienne pas de mesures concrètes sur le foncier. déplorons l’abandon du projet de grande loi foncière dont nous avons besoin pour infléchir les tendances constatées, qui, en l’état, semblent inéluctables. Quels sont vos objectifs en matière d’emplois agricoles, de nombre d’exploitations de surface agricole utilisée (SAU) moyenne ? Je rencontre de nombreux agriculteurs, dans le Gers et ailleurs, qui sont inquiets et n’arrivent plus à se projeter dans un avenir souhaitable pour eux. Ils dissuadent souvent leurs enfants de prendre leur suite… Cela, hélas

une agriculture qui laisse sa place à un modèle agroécologique pleinement inséré dans des territoires ruraux socialement et économiquement vivants ? Devrions nous plutôt chercher une coexistence de ces deux modèles au profit d’un développement territorial assumé

En définitive, et sans préjuger des apports de ce débat, nos attentes relatives à l’approfondissement nécessaire de la transition agroécologique ne sont que très peu, voire pas du tout, prises en compte dans ce texte,

Les Français seront les grands gagnants de cette réussite, tant pour la qualité des productions que la protection de notre biodiversité. La véritable question est donc celle de la compétitivité des agriculteurs français,

Ce défi d’entreprendre est aujourd’hui un casse tête, en agriculture également. Les agriculteurs expriment leur lassitude face à l’avalanche de normes, aux interdictions – responsabilité juridique, installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) –, aux impératifs, parfois complexe – rotation des cultures, jachères, entretien des haies –, et aux accords commerciaux déséquilibrés. La crise agricole de 2023 nous conduit à prendre des mesures qui seront votées définitivement avant le salon de l’agriculture, étape annuelle importante pour les agriculteurs, mais aussi pour les pouvoirs publics, et plébiscité par les Français. Il n’y a pas, d’un côté, le monde agricole et, de l’autre, les défenseurs de l’environnement. L’agriculture, c’est de l’intérêt général, et le Sénat y veille. deux enjeux à cet égard : le vieillissement inédit de la population agricole et le déficit d’attractivité des métiers en agriculture, eu égard au manque de perspectives et aux incertitudes de revenus. de loi d’orientation agricole a été voté en mai 2024 par les députés, à la suite d’une promesse faite par Emmanuel Macron en 2022. Le travail des rapporteurs a permis de clarifier le texte et d’améliorer les outils prévus afin qu’ils soient vraiment au service des agriculteurs.

Les travaux en commission ont conduit à proposer à notre assemblée un principe de non régression agricole, afin que notre souveraineté alimentaire soit protégée au même titre que l’environnement, ainsi qu’un principe de non surtransposition, de manière que la France cesse de pénaliser la compétitivité de son agriculture par un suractivisme normatif.

de la démocratie agricole. Nous sommes donc loin, très loin, de la loi d’orientation de 1962. La commission des affaires économiques a examiné 644 amendements. Le Sénat a donc réalisé un excellent travail de réécriture et de simplification pour améliorer le texte. Je remercie nos deux corapporteurs, Laurent Duplomb,

aussi la volonté d’anticiper la fin d’activité et de promouvoir la formation, la suppression des GFAI, la création d’un guichet unique, la réécriture des dispositions sur les diagnostics modulaires des exploitations, la cartographie des opportunités et risques de marché à vingt

la ministre, mes chers collègues, enfin, nous y voilà ! Malgré l’enlisement qu’a connu ce projet de loi, je tiens à saluer le travail remarquable des rapporteurs, qui ont su transformer un texte initialement peu engageant

la compétitivité et la souveraineté. Ce n’est qu’en renforçant ces deux piliers de notre agriculture que nous pourrons répondre aux défis de l’attractivité et de l’adaptation au changement climatique. L’agriculture française est belle, et bénéficie d’une reconnaissance dans le monde entier. Pourtant, le constat est sans appel : notre agriculture décline. Nous marchons bel et bien sur la tête. La ferme France perd des parts de marché à l’international, tandis que sa production, que l’on a cherché à faire monter en gamme, devient de plus en plus l’apanage d’une minorité de Français aisés. Parallèlement, l’inquiétude grandit face à une agriculture où les fermes familiales laisseraient place à des exploitations industrielles. L’image d’Épinal du paysan de village reste chère au cœur des Français, mais la réalité a évolué la mécanisation a réduit le nombre d’agriculteurs, agrandi les exploitations, et fait de la productivité et de la compétitivité des enjeux incontournables, tout en offrant des conditions de travail bien meilleures. Trop longtemps, ces sujets ont été éludés, comme si l’agriculture ne pouvait être qu’une vocation détachée des réalités économiques et sociétales. Or nos paysans sont avant tout des entrepreneurs, dont l’activité repose sur une logique de coûts et de bénéfices. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille sacrifier tout à la rentabilité. Notre responsabilité est de garantir à nos agriculteurs un revenu digne et d’engager une véritable simplification des normes et des obligations.

Néanmoins, cet article n’est que bavardage s’il ne vient pas concrètement renforcer la protection des agriculteurs face aux trop nombreuses attaques qu’ils subissent. Ces affirmations doivent nous permettre de créer du droit et de défendre concrètement nos agriculteurs. Les mesures du titre II laissent, quant à elles, transparaître une lueur d’espoir en matière d’éducation et de formation des futures générations. Le texte apporte quelques réponses au défi de l’attractivité du métier. En revanche, face au bouleversement démographique à venir, nous allons devoir mieux anticiper la transmission. Le sujet du foncier, véritable marronnier, devra, à cet effet, être au cœur des discussions à venir. Nous avons besoin d’un cap clair pour relancer notre innovation, alléger nos coûts de production et redonner des perspectives à notre agriculture – une véritable loi d’orientation en somme. Madame la ministre, mes chers collègues, alors que nous attendions avec impatience ce texte,… Il faut conclure. … nous pouvons, sur la base du travail de fond mené en commission,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’agriculture française est à un tournant. Vieillissement des exploitants, difficultés d’installation et de transmission, poids administratif écrasant nos agriculteurs demandent des réponses fortes. Ce projet de loi consacre enfin la souveraineté alimentaire comme un intérêt fondamental de la Nation. C’est une avancée nécessaire, mais elle doit s’accompagner d’une programmation pluriannuelle ambitieuse, avec des objectifs précis et des moyens adaptés. Proclamer ne suffit pas, nous devons agir L’un des enjeux majeurs de ce texte concerne l’installation et la transmission des exploitations. Dans le département de la Manche, nous avons recensé 108 installations aidées en 2023 et 96 en 2024. Ces chiffres demeurent cependant insuffisants face aux objectifs affichés par la région Normandie de 450 installations par an, dont 150 dans la Manche. Par ailleurs, l’évolution des modèles d’exploitation doit être prise en compte. En Normandie, terre d’élevage, seulement 38 % des installations concernent l’élevage bovin laitier. Ce constat impose d’adapter nos dispositifs d’accompagnement. Le guichet unique France Services agriculture, désormais rebaptisé France installations transmissions, doit être pleinement opérationnel pour accompagner efficacement ces transitions. Son rôle doit être clair : mettre en relation cédants et repreneurs, et faciliter chaque étape, de l’installation à la transmission. Dans la Manche, entre 2019 et 2024, nous avons perdu 1 100 exploitants agricoles. Certes, cette baisse a été partiellement compensée par une hausse de 1 000 emplois salariés agricoles, mais cela ne suffit pas. Il est impératif d’assurer un renouvellement dynamique et durable des générations agricoles, dont la formation est un élément important. L’article 4 du projet de loi encadre la contractualisation avec l’État, notamment au travers des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) dans l’enseignement agricole. le regrette, mais, malheureusement, depuis 2022, les établissements privés de l’enseignement agricole se retrouvent lésés. L’État a modifié la base de calcul des aides, excluant les financements régionaux qui bénéficient pourtant aux lycées agricoles publics. le manque à gagner est estimé entre 35 millions et 40 millions d’euros, soit 25 % des subventions actuelles. Ce déséquilibre fragilise directement ces établissements et compromet leur capacité à former la prochaine génération d’agriculteurs. Il est impératif de rétablir une égalité de traitement en prenant en compte l’ensemble des financements nécessaires à leur bon fonctionnement. Concernant l’article 13, qui allège la pénalisation de certaines infractions environnementales, nous allons dans la bonne direction. Mais nous devons consacrer un véritable principe de présomption de bonne foi pour nos agriculteurs. Ils ne doivent plus être traités comme des suspects face à des réglementations toujours plus complexes. L’article 14 introduit une nouvelle réglementation des haies, un enjeu fondamental pour nos exploitants. En Normandie, le bocage est un élément structurant de notre paysage agricole. Il est donc essentiel d’accompagner cette transition en prévoyant des dispositifs de soutien technique et financier pour les agriculteurs. La gestion des haies doit être territorialisée afin d’être un atout à la fois pour l’environnement et pour la rentabilité des exploitations. Pour les professionnels de l’agriculture, nous devons veiller à une mise en œuvre équilibrée qui prenne en compte à la fois les exigences environnementales et la réalité du travail des agriculteurs. Enfin, nous devons mieux anticiper les effets des infrastructures électriques et de télécommunications sur les exploitations agricoles. L’amendement que j’ai déposé après l’article 15 vise à imposer un diagnostic préalable obligatoire avant toute installation d’éolienne, de panneaux solaires ou d’antenne relais à proximité d’un élevage.

sur ce sujet important. Ce texte tombe à point nommé, car l’agriculture française, qui fut un fleuron et une fierté nationale, va mal. La profession, dont le travail est dur et souvent peu rémunérateur, n’attire plus les jeunes. La population agricole vieillit. Les mouvements de colère des derniers mois, qui sont toujours latents, nous rappellent cette situation à quelques semaines de l’ouverture du salon de l’agriculture.

Les nombreux territoires agricoles, et notamment le Calvados, ne veulent plus être les variables d’ajustement des politiques publiques. En agriculture, comme pour d’autres sujets, le mot « souveraineté », jadis sacrifié à la loi du marché, s’est imposé à la faveur de la crise du covid 19 et de la guerre en Ukraine.

Les accords commerciaux européens présentés par Bruxelles comme étant exclusivement « gagnant gagnant » posent problème au monde agricole. J’avais eu l’occasion de le souligner, en tant que rapporteur, lors du débat sur le Ceta. Il ne faut pas se voiler la face. Comment défendre notre agriculture quand nos 3 300 milliards d’euros de dette entament notre poids politique et notre crédibilité à Bruxelles ? Quelles marges budgétaires aurons nous dans les prochaines années pour défendre et moderniser ce secteur ? La place importante de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans notre économie est une spécificité partagée par peu d’États européens, d’où notre difficulté à trouver des soutiens. C’est actuellement le cas concernant l’accord avec le Mercosur, que la Commission européenne tente, par divers artifices, de faire avaliser. L’agriculture doit redevenir une priorité. Sinon, nous continuerons à importer toujours plus de produits agricoles, dont certains – on le sait – sont obtenus dans des conditions sociales et environnementales moins bonnes aux nôtres, y compris chez chez nos voisins européens. La France a été le deuxième exportateur mondial de produits agricoles ; depuis lors, nous régressons. Ira t on vraiment vers plus de souveraineté si les jeunes continuent de s’éloigner des filières agricoles, faute d’avenir dans un système de concurrence faussée ? Par solidarité, les Européens ont favorisé les importations ukrainiennes. Résultat, plusieurs filières agricoles ont été déstabilisées. De ce point de vue, la perspective de l’entrée dans l’Union européenne de l’Ukraine, pays qui fut durant des décennies la puissance agricole de l’URSS, est un autre sujet d’inquiétude – il ne faut pas se le cacher – apporter une réponse. La restauration d’une agriculture française compétitive doit être un chantier d’urgence nationale au service de notre souveraineté. Ne commettons pas avec l’agriculture la même erreur funeste qu’avec l’industrie ! C’est une vision de long terme qu’il nous faut, et pas une « politique du chéquier », au coup par coup. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la crise agricole anime la France et la parole publique depuis de nombreuses années. Le sujet est complexe et la crise profonde. Entre 2018 et 2023, le Parlement a examiné pas moins de trois lois Égalim, qui n’ont pas mis fin à la crise et témoignent de l’impuissance politique. Dès 2019, le Sénat alertait pourtant sur l’état de notre agriculture. En 2022, le rapport d’information dénonçait de nouveau la politique anti compétitivité menée par le Gouvernement et appelait à un choc d’ici à 2028. Initialement, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui visait uniquement à répondre à l’urgence du renouvellement des générations. L’urgence est là : la moitié des agriculteurs atteindra l’âge de la retraite entre 2025 et 2026. Or seuls deux départs à la retraite d’agriculteurs sur trois sont remplacés. En septembre 2022, le Président de la République s’engageait à adopter dans les six mois un pacte d’orientation et d’avenir pour notre agriculture portant sur les sujets de l’orientation, de la formation, de la transmission et de la transition. La concertation a été lancée en décembre 2022 et les rapports ont été déposés six mois plus tard. Entretemps, le mouvement agricole de l’hiver 2023 appelait une réponse du Gouvernement. C’est ainsi que le texte issu de la concertation s’est trouvé enrichi de deux titres, l’un relatif à la souveraineté alimentaire, l’autre à la simplification normative en matière environnementale. Ce texte, initialement conçu comme une loi de programmation agricole, a donc été présenté comme une réponse à la crise agricole. Déposé à l’Assemblée nationale en avril 2024, il a été voté le mois suivant, mais il faudra encore attendre neuf mois pour que nous puissions l’examiner. L’instabilité politique a un prix, et ce sont nos concitoyens qui le paient. Devant nos collègues de l’Assemblée nationale, Marc Fesneau, alors ministre de l’agriculture, avait affiché une double ambition : premièrement, « fixer un cap clair lisible aux agriculteurs » ; deuxièmement, adapter nos politiques publiques agricoles afin de relever deux défis immenses et émergents pour notre souveraineté alimentaire. ces ambitions, mais le projet de loi proposé n’est malheureusement pas à la hauteur. Il ne correspond pas à une loi de programmation et ne dresse aucune perspective en matière de revenu, de fiscalité, de foncier et d’innovation. Or la question du revenu est essentielle. Comment penser la transmission si les nouvelles générations ne peuvent vivre de leur travail ? Rappelez vous qu’en 2017 l’une des promesses du candidat Emmanuel Macron était de « permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail ». sept ans que le sujet anime le débat public et que les agriculteurs survivent. Il est temps de répondre à leurs attentes ! Je tiens ici à saluer le travail des rapporteurs et de nos collègues de la commission des affaires économiques, qui ont considérablement enrichi le texte afin de mieux répondre aux ambitions affichées et aux attentes légitimes du monde agricole. Ainsi que l’ont rappelé les rapporteurs, ce projet de loi doit être considéré comme un maillon d’une séquence agricole plus large. En agriculture, comme dans de nombreux autres domaines, la France souffre des effets d’annonce, de l’absence de cohérence des politiques publiques, et encore et surtout de l’absence d’une vision à long et moyen termes. Plus que des belles paroles, les agriculteurs attendent et méritent des avancées concrètes. Dans nos départements, et notamment le mien, la Vienne, les agriculteurs sont en grande souffrance financière et psychologique. Derrière l’agriculture, il y a des femmes, des hommes, des familles qui méritent que nous trouvions enfin les réponses aux difficultés rencontrées,

mérite aussi d’être revisitée à l’aune d’un certain nombre d’études qui ont été faites, notamment dans mon ministère par le CGAAER, sur le poids du foncier dans la reprise agricole.

de redonner un intitulé clair et porteur de sens au titre I. Il s’agit d’aller à l’essentiel, c’est à dire la reconquête de notre souveraineté alimentaire, qui est un impératif.

ne fera de procès d’intention à quiconque dans cet hémicycle ! Nous sommes tous d’ardents défenseurs de nos agriculteurs et de notre agriculture. Il est d’ailleurs arrivé de nombreuses fois que nous nous retrouvions, de façon transpartisane, sur cette ligne de défense, particulièrement au moment de la crise du covid 19 ou lors de la négociation de certains traités de libre échange. Toutefois, l’article 1de ce projet de loi, dans sa rédaction actuelle, définit une orientation beaucoup trop économique et libérale pour que les sénateurs du groupe socialiste puissent en soutenir le principe. En commission, les rapporteurs ont modifié l’intitulé du titre titre I afin que celui ci reflète leurs ambitions, ce qui semble d’ailleurs logique. À notre tour, donc, de le faire ! Nous sommes favorables à la reconquête de notre souveraineté alimentaire – c’est une évidence –, mais nous pensons que celle ci ne saurait advenir à n’importe quel prix, notamment au regard de la préservation de notre environnement et de la sécurité de nos concitoyens. C’est pourquoi,

En évolution (depuis 10 ans), on n’identifie pas de tendance généralisée, notamment pas dans le sens d’une dégradation, même si certaines productions connaissent des évolutions importantes. » Il y a des plus, il y a des moins. Il faut vraiment bien regarder les chiffres, et ne pas en avoir une lecture biaisée. La

à inscrire dans le code rural la définition de la notion de souveraineté alimentaire, et à préciser que la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur. En renforçant nos capacités de production nationales et en protégeant nos agriculteurs de la concurrence déloyale, nous nous assurons que chaque Français ait accès à une alimentation de qualité, tout en consolidant notre indépendance face aux aléas des marchés internationaux. De plus, cet amendement met en avant des mesures concrètes pour atteindre nos objectifs, c’est à dire garantir un revenu décent aux agriculteurs, encadrer les marges abusives des multinationales, renforcer la formation agricole et assurer une politique foncière équitable. Il vise également à corriger un biais réglementaire, en mettant fin aux surtranspositions excessives des règles européennes qui pénalisent notre compétitivité. Enfin, en faisant de la commande publique un levier stratégique, nous privilégions les produits français dans la restauration collective, soutenant ainsi nos filières nationales. Par cet amendement, nous fournissons donc un outil clé pour protéger notre agriculture et assurer un avenir durable à notre souveraineté alimentaire. Quel

L’inscription des notions de « potentiel agricole » dans le champ de protection des intérêts fondamentaux de la Nation et de « non régression de la souveraineté alimentaire soulève de trop nombreuses questions pour voter le texte en l’état. D’une part, nous nous interrogeons sur l’adéquation de ces concepts avec nos engagements environnementaux et avec la nécessité de réaliser un véritable virage agroécologique, que nous appelons de nos vœux. En effet, l’orientation très productiviste que sous tendent ces notions, particulièrement celle d’une « amélioration constante » du « potentiel agricole », rendrait impossible toute décision politique qui n’irait pas uniquement dans le sens d’un accroissement du volume produit. D’autre part, nous considérons comme disproportionné de mettre au même niveau le potentiel agricole, l’indépendance de la Nation, la sûreté nucléaire ou encore la sécurité militaire.

Notre agriculture est confrontée à un défi majeur. La démographie mondiale poursuit sa croissance dynamique, alors que le changement climatique réduit la surface de terres arables. De grandes puissances ont bien compris qu’il existe une géopolitique de l’agriculture : la guerre en Ukraine nous le rappelle tous les jours. La Russie, les États Unis, le Brésil, la Chine et, moins loin de nous, des États en Europe comme la Pologne, l’Italie, l’Allemagne ou les Pays Bas ont repensé repensé leurs politiques agricoles pour relever ce défi. Qu’en est il de la France ? Nos facteurs de production s’étiolent : moins d’hommes et de femmes, en raison du vieillissement de la population moins de terres, en raison de l’artificialisation des sols ; moins d’élevage, en raison de la décapitalisation des cheptels ; moins de moyens de production, en raison de la raréfaction de l’eau dans certaines zones et des solutions culturales pour lutter contre les maladies végétales. le fait que nos dépendances stratégiques sont de plus en plus grandes en matière d’engrais, de protéines végétales, de machinisme, d’énergie, etc. Alors que le monde a sonné la mobilisation générale pour son agriculture, en France, nous continuons à tergiverser. Dans nombre de décisions récentes, les intérêts de la filière n’ont pas été retenus ou, pire encore, ont été totalement ignorés au profit d’autres politiques tout aussi primordiales. À chaque fois, nos résultats agricoles reculent, faute d’être considérés comme une priorité majeure de nos politiques publiques. C’est tout l’enjeu de cette loi

Je vous confirme que ces dispositions permettront une meilleure prise en compte des intérêts agricoles dans la balance des différents intérêts à défendre, tant par l’administration que par le juge, dans une approche au cas par cas. Elles sont la clé pour mieux protéger les moyens de notre souveraineté alimentaire.

respect[a]nt les recommandations du Programme national de l’alimentation et de la nutrition ». En effet, il nous semble indispensable de lier ces deux finalités, de quantité et de qualité, pour accompagner la transition de notre modèle agricole vers davantage de durabilité et d’agroécologie, tout en répondant à des attentes sociétales fortes dans ce domaine. Les deux

un sujet d’intérêt, au même titre que l’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’environnement, le climat, etc. Ce nécessaire rééquilibrage des intérêts en présence est une condition indispensable

de valorisation et de développement appliquées à l’agriculture qui doivent être qualifiées d’intérêt général majeur. La

Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, adoptée en 2018 par l’Assemblée générale des Nations unies, dans laquelle le concept de souveraineté alimentaire

à garantir que la souveraineté s’exerce au bénéfice de l’ensemble de la population en assurant une « alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous

et le renforcement de la biodiversité sont autant de leviers permettant un gain de productivité, ainsi que le maintien et la régénération de la ressource. La biodiversité est un moteur de production. Sans pollinisateurs et autres auxiliaires de cultures, sans matière organique dans les sols et sans diversité des cultures, nous savons qu’aucune productivité n’est possible. L’agriculture joue un rôle crucial crucial dans la préservation de la biodiversité, tout comme, en parallèle, la biodiversité est essentielle aux activités des agriculteurs. Renouer avec des pratiques plus durables est l’ambition même de la transition agroécologique et du Pacte vert européen,

Il s’agit de donner une déclinaison opérationnelle, concrète et collective à la progression de la souveraineté alimentaire de la Nation. Nation. Vous avez tous eu pour ambition de fixer des cibles de production. Ces conférences visent à confier à confier aux filières agricoles, dans leurs différentes composantes, la responsabilité d’établir une stratégie de filière, assortie d’objectifs à horizon de dix ans. Autrement dit, ce n’est pas l’État qui déterminera les objectifs par filière, mais ce sont les filières elles mêmes qui fixeront les modalités, les objectifs et la temporalité de leur progression en matière de souveraineté.

Les premières conférences de la souveraineté alimentaire seraient organisées en 2026, ce qui nous laisse l’année 2025 pour mettre en œuvre ce processus avec les filières. Mesdames, messieurs

pour renforcer les liens entre producteurs et consommateurs. La territorialisation de l’alimentation favorise une agriculture locale, durable et résiliente. Les quatre amendements

cet amendement vise à préciser que le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, présentant une programmation pluriannuelle de l’agriculture française pour les sept années couvrant le prochain cadre financier, doit aussi traiter de l’atteinte des objectifs par mode de production, quand il en existe, comme c’est le cas pour l’agriculture biologique. Cette approche offre la possibilité de mieux suivre la production alimentaire française et de contrôler l’atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement, notamment en matière de développement de l’agriculture biologique.

Cet amendement vise à préciser le contenu du rapport du Gouvernement qui présentera une programmation pluriannuelle de l’agriculture française pour les sept années à venir. À ce stade, ce rapport tend à déterminer les objectifs de production par filière et la stratégie à mettre en œuvre

compris de façon territorialisée. Notre objectif rejoindrait ainsi celui de l’article 2, qui vise une augmentation du nombre d’apprenants d’ici à 2030.

suivie. L’article 1 contient essentiellement des mesures programmatiques, destinées à orienter nos politiques agricoles. Cependant, il contient aussi il contient aussi des mesures que nous jugeons non programmatiques et qui doivent produire des effets juridiques. Or le Conseil constitutionnel nous dit que des dispositions programmatiques et des dispositions normatives ne peuvent pas coexister au sein d’un même article, car cela irait à l’encontre du principe d’intelligibilité de la loi. Cela nous oblige

avancée est la reconnaissance de la souveraineté alimentaire comme intérêt fondamental de la Nation au sens du code pénal, qui est issue d’un amendement de mon collègue Franck Menonville également adopté dans le cadre de la proposition avancée est l’inscription dans le code rural d’un principe de non régression de la souveraineté alimentaire induisant le fait que le potentiel agricole de la Nation ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. Cet apport est issu des travaux de notre commission, et il est majeur.

convient de noter que le Gouvernement fait la même chose au titre II en proposant de supprimer un article du chapitre I pour le déplacer au chapitre II, dans le même objectif d’intelligibilité de la loi.

visent, eux aussi, à réécrire lesdits alinéas en supprimant tout ou partie des trois ajouts cruciaux que je viens d’évoquer. J’y suis donc défavorable.

La problématique que nous avons identifiée lors de nos auditions est que la rédaction de l’Assemblée nationale tend à proclamer des politiques publiques d’intérêt général majeur, en l’espèce la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture. Or une politique publique est, par définition, déjà d’intérêt général. C’est la raison pour laquelle il nous a semblé plus opérant et direct de déclarer l’agriculture d’intérêt général majeur, en tant qu’activité de production. Les syndicats agricoles ne l’ont pas forcément compris, mais je tiens à insister sur ce point.

L’amendement n° 228 rectifié tend à définir la souveraineté alimentaire. C’est intéressant, mais je viens d’indiquer pourquoi ce n’est, à notre sens,

Nous avons travaillé le week end dernier en étroite collaboration avec vous, madame la ministre, pour aboutir à cette rédaction mettant en place une Conférence nationale de la souveraineté alimentaire. La discussion n’a pas été simple ; nous sommes favorables à votre amendement, sous réserve de l’adoption de trois sous amendements, à préciser que, « en amont des négociations du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, le Gouvernement remet au Parlement un rapport

[…] comprend notamment l’élevage, l’aquaculture, le pastoralisme, la viticulture, les semences, l’horticulture, l’apiculture et la sylviculture.

je suis défavorable aux amendements qui ne tiennent pas compte des acquis de l’Assemblée nationale ou de la commission des affaires économiques du Sénat et qui visent à ajouter aux alinéas 1 à 5 des formulations complexes, parfois bavardes, ou des définitions multiples : sécurité sanitaire des aliments, sécurité alimentaire,

Comme vous le savez, la France s’est abstenue sur cette déclaration. Nous sommes attachés à une vision universelle des droits de l’homme, applicables à tous les individus. Enfin, je suis défavorable aux amendements prévoyant que le rapport mentionné à l’article 16 suive spécifiquement les indicateurs de production en matière d’agriculture biologique. Ce suivi existe déjà, en particulier dans le cadre du programme qui repose sur la surveillance de plusieurs indicateurs pour mesurer les progrès et évaluer l’atteinte de ses objectifs. Il ne semble donc pas utile de prévoir dans la loi le suivi d’indicateurs qui sont déjà surveillés annuellement.

Mes chers collègues, avec l’accord de la commission, et compte tenu du nombre de demandes d’explications de vote, je vais lever la séance.